Il appartient aux présidents des CCI de déterminer la meilleure clé de répartition pour assurer la péréquation.

Allonger le délai prévu pour réaliser un don reviendrait à ouvrir un droit à exonération postérieure à la date légale de paiement des droits. Le contribuable devrait alors obtenir une restitution des sommes, ce qui n'est pas praticable. Dans un souci de simplicité, nous souhaitons que le délai pour don sur succession soit maintenu à six mois.

ministre chargé de la ville et du logement, avait lancé un plan national pour inciter les propriétaires de logements vides en zones tendues à les louer. L'objet de cet amendement est de

juin. Quel est l'avis de la commission ?

Le travail qualifié, indispensable pour retrouver le chemin de la croissance, est déjà découragé en France du fait de la très forte progressivité de l'impôt sur le revenu.

comme pour montrer qu'il existerait aujourd'hui en France des marges de manoeuvre pour accroître une pression fiscale déjà record. Ce qu'il n'a pas

! Cette conception punitive de la fiscalité est dangereuse. Elle prive le pays des recettes qu'une fiscalité moins agressive lui apporterait. Elle le prive aussi de retombées économiques liées à la localisation du travail qualifié. On parle On parle souvent d'externalités négatives à propos de la fiscalité écologique ; n'oublions pas les externalités positives liées à la présence des créateurs de richesses et à leur capital humain.

demain. L'intervention publique, c'est une manière de travailler à l'avenir de notre territoire en fournissant les équipements et les infrastructures nécessaires au développement de notre pays et à son attractivité. En 2019, la France était

Ce dispositif n'est pas justifié, le présupposé selon lequel une réduction de la fiscalité sur les dividendes diminuerait le coût du capital supporté par les entreprises n'ayant

L'addition de tous les prélèvements sur le capital y représente 4,4 % du PIB, contre seulement 1,8 % du PIB en moyenne dans les pays de l'OCDE. Moins de capital accumulé, c'est moins d'investissements, moins de richesse, et donc plus de pauvreté.

On raisonne comme si chaque euro gagné avait vocation à être absorbé par l'État. Ce n'est plus à l'État de justifier l'utilité du prélèvement fiscal ; c'est désormais au contribuable de se justifier pour l'argent qu'il a légitimement gagné. Il ne faut pas oublier que l'imposition des revenus épargnés aboutit à taxer deux fois les revenus du travail, déjà touchés fiscalement une première fois au moment de la constitution de l'épargne. On voit donc mal où est le cadeau fiscal, ou même la justice fiscale ! Alors que nous traversons la pire récession depuis 1945, il est plus urgent que jamais, mes chers collègues, de revoir ce rapport à l'impôt. La parole

pas la même chose ! Dans un moment de crise comme celui que nous connaissons, demander un peu de solidarité à ceux qui s'enrichissent en permanence sur le travail,

comme le préconise la Convention citoyenne pour le climat, ce modèle de démocratie dont on ne sait toujours pas exactement ce que compte faire le Président de la République. Par ailleurs, Par ailleurs, les auteurs du présent amendement, estimant que la France est confrontée à un double problème de recherche de nouvelles ressources à la suite de la crise sanitaire et économique et de justice fiscale, proposent de ne pas fixer de montant plancher de dividendes pour l'application de cette hausse de fiscalité.

une fiscalité trop lourde, avec des taux trop élevés, ne peut qu'inciter les contribuables concernés à modifier leurs comportements de façon à échapper, en tout ou partie, au poids de l'impôt. Ainsi a-t-on observé une division par trois, en seulement trois ans, du montant de recettes de cette contribution. Que voulons-nous ? Redistribuer des richesses que l'on ne crée plus ou bien réduire la pauvreté en retrouvant un fort niveau de croissance économique ? Avant de penser à redistribuer les richesses, songeons à les créer. Avant de penser à partager un gâteau qui s'est amenuisé, songeons à le reconstituer et à lui rendre sa taille d'avant le coronavirus. Pénaliser fiscalement ceux qui ont, par le passé, fait la preuve de leur capacité à entreprendre, à investir, à innover pénalisera au bout du compte l'ensemble des Français, en freinant le redémarrage de notre économie.

du 14 juillet, le chef de l'État a assuré que les deux années de fin de mandat seraient consacrées à la relance et à l'emploi. Cette période exceptionnelle étant une opportunité pour la France de se réinventer, nous proposons de réinventer également notre modèle fiscal. pays est, en apparence, celui dont la fiscalité est la plus importante, en réalité, entre les multiples déductions, exonérations, abattements ou autres portes de sortie, les filets laissent passer les grosses fortunes et il ne reste finalement que les contribuables qui ne sont pas forcément les plus riches.

De la même manière, celles et ceux qui ont la chance de gagner plus de 500 000 euros par an doivent actuellement s'acquitter d'une contribution exceptionnelle de 4 % ; nous proposons de la rehausser pour la fixer à 10 %. L'objectif est avant tout d'instaurer une solidarité entre les plus aisés et les plus précaires. La crise sanitaire a démontré la nécessité d'un système de protection sociale de qualité ; par conséquent, il convient de taxer les revenus les plus importants pour financer les politiques publiques en faveur de la relance économique, sociale et écologique.

Pas sûr ... Évidemment, M. Cadic aura un peu de mal, je peux le comprendre, mais, après tout, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que nous soyons unanimes pour saluer cette innovation de Nicolas Sarkozy,

un élément qui n'est pas de nature à restaurer la confiance. Pour que nos concitoyens investissent et consomment, il faut que les règles soient stables. Ce raisonnement me conduit

de participer à la baisse du chômage, avant la crise du covid. C'est une politique que nous voulons poursuivre en cette période de sortie- espérons-le -de crise. La stabilité de cette trajectoire est importante pour nous. De la même manière, nous considérons qu'il existe des outils de financement de la solidarité- M. Karoutchi en rappelait la genèse de 2012 -, notamment la contribution sur les hauts revenus, qui permet d'embrasser les revenus au-delà des seuls revenus salariés.

aux Américains beaucoup moins important, en tout cas pour les moins favorisés. C'est un élément important à prendre en compte. En outre, je veux aussi rappeler le rôle économique de l'État dans la création de richesse. L'État n'est pas un puits sans fond, les dépenses réalisées

nous ferons une grande table ronde pour remettre à plat l'ensemble de la fiscalité française, de manière à enfin trouver des solutions ». Il ne l'a jamais faite

Il se trouve que notre pays est en situation de péril ; il s'agit de trouver des mesures qui soient acceptables par une grande majorité de la population. Soumettons-lui ces mesures ! On a

Voilà ce qui n'est plus acceptable, ce qui n'est plus accepté : la part des impôts les plus injustes dans les recettes fiscales de l'État, car, ce que finance l'État, ce sont les services publics qui doivent contribuer à la redistribution. Or cette redistribution, même si c'est l'une des meilleures au monde,

pendant la période. Il s'agit d'une contribution sur l'augmentation des résultats d'exploitation par rapport à la moyenne des trois dernières années, correspondant à 80 % de l'augmentation de ce résultat. J'ai pérennisé le dispositif,

nous avons recensé 1,9 milliard d'euros de gestes commerciaux consentis par les sociétés d'assurances à leurs assurés et la Fédération française de l'assurance pilote un plan d'investissement au profit des PME et des TPE à hauteur de 1,5 milliard d'euros. C'est un engagement

fort des chiffres que nous aurons eus. Monsieur le rapporteur, vous n'avez pas qualifié le travail de mon groupe pour améliorer ce dispositif. Vous avez dit que c'était compliqué. Nous proposons un dispositif très simple-

qui devait être rendu aurait évidemment éclairé le débat ... Le Sénat avait voté le rétablissement d'une taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l'assurance, mise en place durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, en 2011. Il s'agissait évidemment de prendre en charge les pertes d'exploitation pour le secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques. Cet amendement avait été voté dans le cadre du PLFR

vous ne voulez pas de taxe, proposez-nous un mécanisme qui corrige cette situation ! Nous appelons à la modération des dividendes.

dans l'objet de l'amendement de Mme Férat : il y est écrit que celui-ci « propose de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l'assurance, mise en place en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy »-

les collectivités territoriales, notamment les régions, et les assurances. Nous étions toutes et tous d'accord, lors du premier budget rectificatif, pour dire que les assurances ne jouaient pas le jeu.

1,5 milliard de financements en fonds propres en direction des TPE-PME, notamment pour le secteur médical et les start-up.

Il arrive de signer des amendements par amitié et de les retirer par conviction ... C'est exactement ce que je fais

à la rentrée prochaine. Le PLF pour 2021 que nous préparons instaure une première diminution de la taxe d'habitation pour les 20 % des contribuables restants. Nous allons donc vers l'extinction de la taxe d'habitation, raison pour laquelle nous préférons maintenir le dispositif de compensation, tel qu'il existe, pour l'exonération « vieux parents » que créer de manière très temporaire

En outre, la légitimité même de ce dispositif, qui nous semble coûteux pour la puissance publique, peut être remise en cause. Nous vous engageons à supprimer cette disposition malvenue de l'Assemblée nationale.

d'épargne avaient été utilisés pour être injectés dans l'économie, grâce à un dispositif de nature comparable. Nous n'avons pas d'opposition de principe sur l'article 4. Nous souhaitons, au contraire,

l'avis du Gouvernement ? La disposition adoptée par l'Assemblée nationale permet d'exonérer les dons au sein d'une même famille, quand ces derniers sont consacrés à la création ou au développement d'une entreprise de moins de 50 salariés.

voulons étendre le champ des dépenses éligibles aux opérations de rénovation énergétique, d'acquisition et de construction de la résidence principale. Nous avons donc à la fois vérifié la compatibilité avec le régime des aides d'État

à compléter le débat, madame la présidente. Sur la question de la définition des liens familiaux, nous renvoyons au droit commun. M. Raynal me pardonnera une seconde fois ma malice, mais, dans la proposition de loi du groupe socialiste et républicain

afin d'orienter l'épargne des Français vers le financement des associations et des TPE-PME dans les domaines de la transition écologique, de la sécurité sanitaire et de l'innovation sociale. plaire -l'une des quarante-cinq propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le parti socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier-

: La parole est à M. Maurice Antiste. Mise en place en France par la loi de finances pour 2012, la taxe sur les transactions financières est une taxe boursière s'appliquant sur les actions des sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros. à l'origine à 0,1 %, le taux de taxation est actuellement de 0,3 % de la valeur d'acquisition. Elle a été instaurée pour répondre à un triple objectif : solliciter la contribution du secteur financier pour redresser les finances publiques ; réguler le marché boursier ; demander l'adhésion des autres États membres de l'Union européenne pour une portée plus générale de la taxe.

450 millions affectés au budget de l'État et 533 millions à l'aide au développement. En 2017, avec l'augmentation du taux à 0,2 %, le rendement s'élevait à 1,45 milliard dont 652 millions affectés au budget de l'État et 798 millions à l'aide au développement. Cet amendement vise donc à augmenter la taxe sur les transactions financières pour la porter au taux de 0,6 %, ainsi qu'à élargir son assiette aux transactions intrajournalières, c'est-à-dire les achats et ventes de titres réalisés au cours d'une même journée à des fins spéculatives, comme le prévoyait la loi de finances pour 2017 avant l'abrogation de cette disposition dans la loi de finances pour 2018.

leurs projets d'investissement. Aussi, l'obligation qui leur est faite de disposer d'au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit pour ouvrir droit à un avantage fiscal pour les souscripteurs sera, pour certaines d'entre elles, impossible à réaliser, sauf à engager artificiellement leurs fonds à cet effet, et souvent au péril du devenir de la société. Cet amendement vise à décaler d'un an cette obligation afin de ne pas pénaliser les investisseurs dans les sociétés nouvelles, en tenant compte de la période d'au

de voir leurs déductions non autorisées. Il s'agit en général de petits porteurs qui entrent dans le capital de sociétés et qui n'ont pu voir le projet aboutir dans les temps impartis- il s'agit

En revanche, l'amendement déposé chaque année par le président Éblé est bien mieux rédigé puisqu'il exonère de CSG et d'imposition le loto du patrimoine,

sont assurés d'obtenir une recette au moins égale à celle qu'ils percevront en 2020 pour la TFPB : la loi de finances pour 2020 dispose explicitement que le montant versé aux départements en TVA sera égal non pas à un pourcentage de la TVA perçue en 2021, mais à la somme perçue en 2020.

Une précision supplémentaire, madame la présidente : j'ai un souvenir assez exact du débat que nous avons eu sur les mécanismes de garantie. La loi de finances pour 2020 prévoit, sur l'initiative du Gouvernement, un mécanisme de garantie en vertu

celui de l'année précédente. Si je puis me permettre une expression un peu triviale, nous avons prévu une forme de « ceinture de sécurité » ; M. le rapporteur général voulait, lui, que ce soit ceinture et bretelles, ce qui nous paraissait peut-être un peu excessif et nous engageait un peu trop. La parole

Je rappelle que la suppression de la TH entraîne de fait une modification de ces potentiels, et donc de tout ce qui en découle, c'est-à-dire de tous les systèmes de répartition entre collectivités locales,

Je vous interroge donc, monsieur le ministre, sur notre capacité à avancer de manière sérieuse pour, dans un premier temps et, neutraliser cet effet

Dernier élément pour vous rassurer, monsieur Raynal : l'effet de la réforme de la taxe d'habitation sur le calcul des PFiA et, éventuellement, sur les modalités de calcul des dotations n'interviendra pas avant 2022, puisque le PFiA qui intégrera le nouveau panier fiscal sera celui de 2022, calculé sur les éléments connus de 2021, ce qui nous laisse quelques mois, là encore, pour ajuster le tir autant que nécessaire- je redis là ce que j'avais dit en décembre dernier ici même devant vous.

du budget de l'État au profit des collectivités territoriales, qui représentent- on le voit en loi de finances chaque année -des sommes importantes : largement plus de 40 milliards d'euros.

et tarifaires qu'essuient les collectivités sont estimées à 7,4 milliards d'euros par la mission gouvernementale sur l'impact du covid-19 sur les finances locales. Pour le bloc communal, les pertes sont estimées à 2,5 milliards d'euros.

du reste. Pour avoir beaucoup échangé avec la présidente de la région et avec les services d'Île-de-France Mobilités, je pense que la vérité se situe entre la proposition du Gouvernement et la demande de la présidente de la région. Le Gouvernement devrait être un peu plus ouvert, parce que

proposons, par cet amendement, de créer deux prélèvements et de déterminer les modalités de calcul des dotations individuelles par collectivité. Le premier de ces prélèvements sur recettes de l'État permettrait d'accompagner les collectivités locales qui perdent des ressources importantes, et donc de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne 2017-2019. Le deuxième prélèvement leur permettrait

La difficulté que pose cet amendement est qu'il mélange deux choses : une approche par les recettes et une approche par les coûts. Autant je suis favorable à la compensation des pertes de recettes, autant je considère que l'approche par les coûts est assez dangereuse, et même contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à la réécriture totale de l'article 5. En revanche, la commission a essayé d'améliorer

Le Gouvernement a fait le choix de créer un dispositif de garantie de recettes, et je tiens à souligner que ce dispositif est absolument inédit. Lors de la dernière crise systémique de 2008-2009, le seul outil qui avait été mis en place en matière de recettes pour les collectivités était la possibilité de bénéficier d'une avance d'une annuité sur la section d'investissement. Mais aucun dispositif n'avait été mis oeuvre pour compenser la perte de recettes, au niveau du bloc local comme au niveau du bloc départemental, avec deux années consécutives de baisse très forte des DMTO.

les collectivités restent totalement autonomes dans leur fonctionnement- et c'est heureux ! Nous leur apportons une sécurité, mais nous n'entrons pas dans une logique de compensation de dépenses. L'amendement de M. Marie présenté par M. Joly vise à proposer une compensation des pertes de recettes tarifaires. Nous ne sommes pas entrés sur ce

Quant au déficit prévisionnel de la sécurité sociale, il s'élève à 50 milliards d'euros. Autrement dit, les trois blocs de dépenses publiques, affaires sociales, État, collectivités, sont évidemment mis en difficulté par la crise que nous connaissons, et je crains qu'hélas aucun des blocs n'en sorte totalement indemne. des recettes tarifaires, nous avons en vue une autre difficulté, qui explique que nous ne les ayons pas prises en compte : c'est souvent sur les services engendrant des recettes tarifaires que nous observons des économies de constatation, qui sont par nature difficiles à évaluer, et nous ne sommes pas entrés dans cette logique-là.

de le défendre. Avec l'arrêt de l'activité durant le confinement et plus largement pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, les collectivités- nous l'avons dit à de multiples reprises -ont perdu une partie importante des recettes tarifaires de leurs services publics locaux. Le phénomène est particulièrement marqué pour ce qui concerne les activités dites touristiques- camping municipaux, gîtes communaux, établissements thermaux, etc. -, pour lesquelles les pertes de recettes tarifaires sont quasi totales du fait de la fermeture des sites. À l'instar de ce que le présent projet de loi prévoit pour les communes et leurs groupements, cet amendement vise à rendre éligibles au mécanisme de compensation des pertes de recettes tarifaires engendrées par la crise du coronavirus les régies municipales qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) touristique. Quel est l'avis de

avec une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire lorsque les droits de mutation auront retrouvé un niveau équivalent au niveau antérieur. À ce moment-là, les départements seront en mesure de rembourser l'avance qui leur a été consentie. Vous le voyez, nous ne négligeons pas la situation des départements,

que l'essentiel de leur financement était lié à des recettes d'activité, et non pas à des subventions d'origine publique. Nous avons aussi tenu compte d'une autre différence pour les services en régie directe, dans la mesure où, en 2020, les collectivités, tant par les mécanismes de garantie de ressources que par le maintien des dotations de fonctionnement, ont vu leurs ressources de fonctionnement relativement bien préservées. Cela permet d'assurer le même niveau de financement pour tout ce qui relève d'une gestion en régie directe. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas entrés dans un dispositif de compensation,

J'en profite pour revenir sur un sujet qui va être prégnant et qui concerne justement ces redevances d'occupation du domaine public : le stationnement. Dans les EPT du territoire de la métropole du Grand Paris, on va subir un écroulement des recettes de stationnement en 2020, alors même que les

C'est ce qui a amené le Gouvernement à donner un avis défavorable à cet amendement, considérant que les difficultés que vous soulignez sont assez largement surmontables. Je le disais voilà un instant en réponse à

Quand on a mis en place la métropole du Grand Paris, j'ai quelques souvenirs de débats héroïques. N'est-ce pas, Philippe ? Ces établissements publics territoriaux étaient des extraterrestres.

au moment de la mise en place de la métropole. Ne venez pas, après, nous en faire le reproche. Nous avons nous aussi des pertes lourdes, comme les autres ; les autres sont compensés, mais pas nous, parce que vous nous avez imposé un statut que nous ne voulions pas au départ, mais qui arrangeait le Gouvernement pour ses strates.

C'est juste une question d'égalité de traitement. Je comprends que ces ovnis juridiques que sont les EPT soient souvent oubliés quand il y a de nouvelles dispositions,

Mme Muriel Cabaret. Cet article prévoit d'instituer une dotation versée par l'État afin de compenser pour les communes et les EPCI à fiscalité propre une partie de la perte de leurs recettes fiscales et domaniales.

Il est prévu que ce dispositif de compensation s'applique à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE), la rédaction de cet article précisant que la part de la dotation attribuée à une commune ou à un EPCI à fiscalité propre est égale à la différence entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020. En revanche, les syndicats intercommunaux qui perçoivent la TCCFE ne pourront pas bénéficier de ce dispositif, qui vise uniquement les communes et les EPCI à fiscalité propre.

pour accompagner financièrement le bloc communal, à savoir les communes et les EPCI à fiscalité propre, qui connaissent des pertes de recettes fiscales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire.